Nul n'est obligé de s'engager dans la fonction publique. De moins en moins d'ailleurs, aurais-je tendance à dire, puisque, au terme des dispositions qui ont été adoptées, il n'est il n'est même plus nécessaire d'être titulaire pour exercer. Cela étant dit, le pantouflage, le rétropantouflage et leurs excès sont les mamelles qui alimentent les procès faits aux élites,

en prohibant toute mise en disponibilité pour convenances personnelles avant le terme de cette période de quinze ans ; en généralisant l'obligation de remboursement en cas de rupture anticipée de cet engagement de servir ; en confiant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, la mise en oeuvre de la procédure de remboursement.

au terme de leur formation rémunérée. En effet, faute de procédure de recouvrement clairement définie et de centralisation de la mission de recouvrement, il semblerait que cette obligation soit mise en oeuvre de façon très disparate, en cas de départ anticipé de la fonction publique, selon le corps d'origine. d'origine. Nous proposons, par cet amendement, de renforcer les dispositions légales, afin de contraindre chaque administration à se saisir de ce problème. madame la présidente. la somme qu'un ancien élève d'une école de la haute fonction publique doit rembourser, lorsqu'il résilie avant terme son obligation de servir dix ans l'État qui a financé sa formation et l'a rémunéré pendant cette période. On connaît de nombreux exemples de ces pratiques qui conduisent de jeunes hauts fonctionnaires, dont l'ascension a été permise par l'État, à quitter l'administration publique pour aller pantoufler dans de grandes entreprises privées, en espérant de plus grasses rétributions. À son corps défendant, l'État a donc formé en son sein de futurs cadres stratégiques ou dirigeants du secteur privé qui défendront ensuite, et parfois contre lui, des intérêts financiers contre l'intérêt général. À cette pratique condamnable s'ajoute celle du rétropantouflage : un ancien haut fonctionnaire passé au privé revient dans la haute fonction publique. Ces allers-retours suscitent un trouble sérieux dans l'opinion quant à l'action d'une partie de la haute administration,

d'une simplification utile. Ces amendements ayant été rectifiés à la demande de la commission, ce dont je remercie leurs auteurs, la commission émet un avis favorable. L'amendement n° 253 est satisfait par le droit en vigueur : le remboursement de la pantoufle est d'ores et déjà L'avis est donc défavorable.

des anciens élèves de l'École nationale d'administration, qui s'applique par homologie à une soixantaine de corps de fonctionnaires de la fonction publique d'État, permet l'établissement d'un titre de perception avec un caractère exécutoire. Ces amendements identiques étant satisfaits par le droit existant, l'avis

En effet, nous disposons actuellement de bien peu de données sur la question. Mais cette demande s'est perdue dans les méandres législatifs. Cet amendement vise à réitérer cette demande, car un tel rapport permettrait également d'amorcer une réflexion au sein de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, en vue d'une harmonisation des régimes de recouvrement de la pantoufle entre les corps.

Cet amendement a pour objectif de lutter contre les conflits d'intérêts dans la fonction publique, en interdisant à tout ancien fonctionnaire ou agent public d'exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. Il interdit également à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée, ou pour une société de conseil, d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liées aux secteurs d'activité dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. Nous considérons que cette mesure est tout à fait indispensable, particulièrement dans le cadre de ce projet de loi qui accentue la contractualisation de la fonction publique, ce qui aura inévitablement pour effet d'entraîner une confusion entre les intérêts publics et privés. Cet effet est déjà à l'oeuvre avec le pantouflage, lequel crée un phénomène de porosité entre les élites administratives et les élites économiques, ce qui nuit gravement

Un millier de fonctionnaires d'État seraient concernés chaque année par le pantouflage, c'est-à-dire par le fait de passer du secteur public au secteur privé. Jadis pratiqué en fin de carrière, ce système s'est généralisé et les risques de conflit d'intérêts n'ont ainsi jamais été aussi nombreux. Par ailleurs, le pantouflage fonctionne aussi dans l'autre sens le rétropantouflage. De plus en plus de hauts fonctionnaires partis dans le privé reviennent vers le public. Il s'agit d'un problème structurel à notre pays, qui est le seul à connaître une telle perméabilité entre les intérêts privés et les intérêts publics. L'Organisation s'en est inquiétée il y a quelques années dans un rapport. Selon elle, « les relations proches entre, d'un côté, les régulateurs et le pouvoir politique et, de l'autre, l'industrie de la finance et ses lobbyistes, sont alimentées par le recyclage régulier de personnel entre ces deux univers » et « s'attaquer aux portes tournantes constitue le début d'un processus indispensable afin de restaurer la confiance des citoyens dans le système politique et le fonctionnement des marchés financiers ». Quel est l'avis de la commission ? Ces amendements

Ces amendements me semblent en grande partie satisfaits par l'article 16 AA, que nous avons adopté en commission sur l'initiative de leurs auteurs, interdisant, pendant trois ans, à un fonctionnaire d'exercer une fonction de représentant d'intérêts auprès de son ancienne administration. Les avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves qui seront émis par la HATVP vont dans le même sens. À l'article 16, nous avons d'ailleurs substantiellement renforcé la portée de ces avis. En outre, les termes employés dans les amendements, notamment sur les liens « directs

ainsi libellé : La parole est à M. Jérôme Durain. Nous proposons, au travers de cet amendement, de mettre un terme à un type de pantouflage qui, depuis la crise financière de 2008, laisse planer un doute sur l'impartialité d'une partie des hauts cadres de la fonction publique. On ne peut être chargé de surveiller un système bancaire qui a créé une des plus grandes crises depuis celle de 1929 et envisager de poursuivre sa carrière professionnelle dans une des banques faisant l'objet de cette surveillance. On ne peut conseiller les décideurs politiques sur les conséquences de la mise en oeuvre de contraintes supplémentaires en matière de gestion du risque systémique du secteur bancaire et penser pouvoir aider ultérieurement une banque à s'émanciper de ces contraintes. On ne peut mettre en oeuvre la surveillance fiscale des flux financiers et imaginer conseiller, dans le futur, une des institutions surveillées. En clair, nous devons définitivement lever le doute sur l'impartialité de hauts fonctionnaires du ministère des finances qui pourraient envisager de monnayer leurs compétences dans un secteur d'activité qui reste un secteur à risque pour notre économie.

y a mille raisons, au moins une en tout cas, de faire un sort particulier aux inspecteurs des finances : ils pantouflent à 70

-pour le service public. Mais je crois que ce qui se passe précisément à la direction des finances pose légèrement problème. M. le secrétaire d'État. Au risque d'être insistant, monsieur le sénateur, la « direction des finances » n'existe pas. Nous avons une direction générale des finances publiques, au sein de laquelle il y a une direction de la législation fiscale, et une inspection générale des finances, qui est considérée comme un grand corps. corps. Il serait utile, pour nourrir votre argumentation, que je vous remette, à l'occasion de la prochaine séance, un organigramme complet des services du ministère de l'action et des comptes publics, ainsi que du ministère de l'économie et des finances. de colère, parce que- je le répète -à la place qui est la mienne aujourd'hui, je peux témoigner de la qualité de ces hommes et ces femmes, et de celle de leur engagement. La France et les représentants du peuple français devraient s'enorgueillir d'avoir une haute fonction publique et, au-delà,

qui est sanctionné par le code pénal, et de trafic d'influence qui est, lui aussi, sanctionné par le code pénal.

Cet amendement serait également plus sévère pour les élus locaux, alors même que la définition de la prise illégale d'intérêts pose un véritable problème. En ce qui concerne les mobilités du privé vers le public, je rappelle que nous avons amélioré,

et pour assurer la quiétude de ces braves gens qui se dévouent, de prévoir un délai suffisant pour que ces derniers ne soient pas soumis à la tentation.

Nous vivons aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une forme de crise démocratique. Nombre de nos concitoyens, souvent poussés par des forces que

d'abord, de la communication par le président de la HATVP « des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d'une déclaration d'intérêts et d'activités, d'une déclaration d'intérêts ou d'une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ces instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d'intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement celui-ci ». Il s'agit, ensuite, de la communication par l'administration fiscale « d'une attestation constatant qu'à la date de la demande et en l'état des informations dont dispose cette administration,

? Dans la loi pour la confiance dans la vie politique, le Sénat a créé, sur l'initiative du président Bas, une procédure de contrôle avant la nomination des membres du Gouvernement. Le Président de la République peut désormais consulter la HATVP, l'administration fiscale et le bulletin n° 2 du casier judiciaire. L'amendement de M. Durain propose d'étendre cette procédure aux nominations au titre de l'article 13 de la Constitution et à certains emplois publics. La commission des lois y est défavorable, pour deux raisons. D'abord, parce que l'amendement nous semble largement satisfait pour les emplois publics : les personnes concernées doivent remplir une déclaration d'intérêts en amont de leur nomination. Il en va de même pour le casier judiciaire qui doit être vierge. concernant les nominations au titre de l'article 13 de la Constitution, qui semblent d'ailleurs éloignées du champ du projet de loi, les éventuelles révisions institutionnelles seront l'occasion de renforcer les pouvoirs du Parlement. Quel est l'avis du Gouvernement

et supprimés par l'Assemblée nationale, relatifs à la déontologie de la haute fonction publique. Il s'agit en l'occurrence d'un amendement de Marie-Noëlle Lienemann qui interdisait de nommer à une fonction d'intérêt général relevant de la procédure de l'article 13 de la Constitution une personne qui aurait travaillé, au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ayant des liens avec l'organisme au sein duquel elle exercera sa fonction. Par ailleurs, cet article interdit la participation des personnes exerçant actuellement une fonction d'intérêt général à une délibération concernant une entreprise dans laquelle elles ont travaillé au cours des trois années précédant cette délibération et qui entretient des liens avec l'organisme auquel elles sont rattachées.

La procédure de l'article 13 dépasse très largement le champ du projet de loi. Elle pourrait d'ailleurs être renforcée à l'occasion des prochaines réformes institutionnelles. Par ailleurs, les auditions devant les commissions parlementaires permettent de prévenir les conflits d'intérêts. De plus, l'adoption de cet amendement empêcherait, par exemple, la nomination à la tête de la Caisse des dépôts et consignations d'une personne ayant auparavant dirigé une de ses filiales. Nous serions alors contraints de prendre un fonctionnaire de Bercy, ce qui n'est sans doute pas l'intention des auteurs de l'amendement. La situation est identique pour l'Autorité de sûreté nucléaire. Nous avons besoin de spécialistes pour un certain nombre de postes sensibles. Il s'agit de ne pas bloquer des évolutions de carrière ou des nominations qui pourraient être tout à fait pertinentes, en vertu d'un principe qui se retournerait contre la volonté du législateur. Enfin, les organismes concernés possèdent déjà

l'avis du Gouvernement ? Les occasions pour le Gouvernement d'être totalement d'accord avec le président Philippe Bas sont trop rares à mes yeux. Je saisis l'occasion pour le conforter sur ce point ! J'ajoute que les emplois ciblés dans cet amendement

Ce qui se passe réellement, c'est qu'on a abattu progressivement les barrières entre le public et le privé, et on passe de l'un à l'autre

est d'accord. En effet, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait prévu personne exerçant une fonction dans le privé pouvait continuer à bénéficier des avantages du statut de la fonction publique : l'avancement, le droit à la retraite, etc. Mais où va-t-on ?

d'État- c'est dire ! - et à rétablir un minimum de séparation entre l'exercice des prérogatives publiques et l'exercice d'un métier privé.

de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, un fonctionnaire placé en disponibilité pour exercer des fonctions professionnelles dans le secteur privé conserve ses droits à avancement et à retraite.

l'avis du Gouvernement ? La mesure visée ici est une disposition de la loi du 5 septembre 2018 qui, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, vise, d'une certaine manière, à aligner, en termes de droits pour les agents, le régime de la disponibilité pour convenances personnelles sur celui du détachement.

En réalité, nous l'avons pensée comme une modalité tendant à faciliter les retours dans la fonction publique d'agents publics faisant valoir leur droit à une disponibilité. Nous avons aujourd'hui des agents publics-

acquise pendant cette période peut être extrêmement bénéfique à l'administration publique. Je prends un exemple volontairement caricatural : si un agent des services fiscaux

à faciliter le retour dans le public d'agents qui ont vécu une expérience dans le privé et, ensuite, à protéger le déroulement de carrière d'agents et d'agentes qui n'ont pas fait le choix d'une disponibilité, mais qui la subissent. J'ajoute pour compléter mon propos

sont ceux pour lesquels le pantouflage est une modalité d'exécution de leur carrière. Ils ne perdent rien

Cela me fait penser à ce que disait un ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre : « Les banques prospèrent à l'international et viennent mourir au pays.

je devais être promue. Du jour au lendemain, on a stoppé ma promotion ; quand je reviendrai, je retournerai tout en bas, ce qui posera un véritable problème. Aujourd'hui, en l'état actuel, je pourrais difficilement retourner dans la fonction publique, même si c'était mon choix. Moi aussi ! Si cette disposition s'applique aux mandats des élus, c'est très bien ; si ce n'est pas le cas, il faudrait peut-être y penser. Je ne pense pas que quelqu'un

et a de meilleures relations avec ses administrés ou avec ses interlocuteurs que sont les élus qui lui succéderont pour mettre en oeuvre des politiques publiques. Je soutiens complètement cette disposition, d'ailleurs validée par le Conseil d'État, puisque le décret a été publié au mois de mars dernier.

qui n'est pas accompagnée, malgré le décret pris le 27 mars 2019, du maintien du déroulement de carrière et des dispositions visées par la loi du 5 septembre 2018. Je rejoins

que certaines demandes de disponibilité pour convenances personnelles ne sont pas choisies, lorsqu'elles accompagnent un mouvement de mutation d'office, elles sont toujours soumises à un accord de la hiérarchie,

Quand on examine le parcours des pantouflards professionnels, on s'aperçoit qu'il y a deux voies

réduire la fréquence avec laquelle les membres de cabinets peuvent pantoufler, ce ne sera pas plus mal.

les nominations au tour extérieur sont déjà encadrées. À titre d'exemple, le vice-président du Conseil d'État émet, sur chaque projet de nomination, un avis qui prend en compte les fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, son expérience et les besoins du corps ; le sens de cet avis est d'ailleurs rendu public.

En effet, une interdiction générale et absolue d'exercice d'une activité de représentant d'intérêts, sans limitation relative à son champ d'application matériel, serait, à nos yeux, contraire à la Constitution. Par ailleurs, les dispositions relatives au départ vers le secteur concurrentiel, notamment en vue d'exercer des activités de conseil, telles qu'elles sont prévues par les articles 25 et 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, permettent déjà d'encadrer ce type de situations, tout comme les dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite la suppression de cet article.

Cet article prévoit que, pendant une durée de trois ans, les anciens fonctionnaires s'abstiennent d'exercer une fonction de représentant d'intérêts auprès de leur ancienne administration. Il ne s'agit pas d'une interdiction générale et absolue. En effet, l'intéressé pourra toujours exercer des activités de lobbying ; seulement, il ne pourra

La communication de données portant sur des éléments de rémunération doit viser un but précis et s'inscrire dans un cadre qu'il convient de définir. Ainsi, si la volonté de récolter des informations portant sur les rémunérations à des fins statistiques, comme le précise l'alinéa 2 du présent article, s'entend tout à fait, je m'interroge sur l'intérêt de leur publication sur le site internet des collectivités et des administrations concernées. Dans un contexte national déjà sensible, la pertinence et la justesse des conclusions qui peuvent être tirées par les internautes de la publication de tels éléments peuvent être mises en cause. C'est pourquoi je propose la suppression de cet alinéa.

de ces dix rémunérations. En outre, je le rappelle, la commission d'enquête sénatoriale sur la haute fonction publique a appelé à plus de transparence en la matière.

nos amendements sur ce thème, vise à inscrire dans l'annexe du rapport annuel sur l'état de la fonction publique, remis par le Gouvernement au Parlement, des éléments de nature à favoriser un meilleur contrôle des dispositifs de remboursement de la pantoufle des hauts fonctionnaires.

outre, les informations publiées concerneront également des rémunérations inférieures à 120 000 euros bruts annuels, donc l'amendement n° 245 pourrait restreindre le contenu du rapport du Gouvernement, ce qui ne semble pas souhaitable.

second lieu, les autorités administratives indépendantes, auxquelles il faudrait d'ailleurs ajouter les autorités publiques indépendantes, sont régies par un statut spécifique, d'origine sénatoriale. Ce statut leur garantit une liberté de recrutement, dans les limites de leur budget et,

près de 800 000 salariés -, comme Areva, ont besoin de compétences pointues, surtout dans des domaines concurrentiels ou qui vont le devenir. Surtout, les fonctionnaires qui travaillent dans ces structures seraient défavorisés par rapport aux agents de droit privé,

au moment de sa nomination ou de son renouvellement ; il s'agit là de la rédaction issue de l'Assemblée nationale. Ce dispositif s'inspire du droit applicable aux présidents de conseil d'administration et aux directeurs des établissements publics de l'État.

territoriale, la MNT, 91 % des agents et 75 % des élus sont favorables à l'amélioration de la protection sociale des agents. Malheureusement, vous avez refusé, monsieur le secrétaire d'État, d'inscrire dans la loi le principe de la participation obligatoire. Pourtant, dans le secteur privé, les employeurs sont obligés de participer au financement de la protection sociale complémentaire des salariés. Le Gouvernement, qui mène par ailleurs une politique d'affaiblissement du périmètre de la sécurité sociale au profit des complémentaires privées, refuse donc aux agents publics de pouvoir se soigner dans de bonnes conditions. Le Gouvernement doit, d'une part, acter la participation obligatoire au financement de la protection sociale complémentaire avec un minimum de 50 % et, d'autre part, garantir aux collectivités territoriales une dotation de l'État fléchée pour améliorer la prise en charge de la santé et la prévoyance des agents. Cette mesure n'est pas portée uniquement par notre groupe, puisque, selon un sondage IFOP-MNT d'octobre 2017, les décideurs territoriaux sont favorables à 75 obligatoire de la participation financière des collectivités à la protection sociale des agents, avec au moins 15 euros en santé par mois et par agent et 5 euros en prévoyance. L'article 17 renvoie aux ordonnances et aux négociations avec les organisations syndicales, alors que le bon sens aurait voulu

Je rappelle que 67 % des agents publics ressentent des douleurs physiques liées à leur position de travail, et 35 % ont le sentiment que leur travail dégrade leur santé. Le vieillissement des effectifs renforce cet enjeu, les agents de 50 ans et plus représentant aujourd'hui 33,4 % des effectifs des effectifs de la fonction publique, avec un vieillissement encore plus marqué dans le versant territorial, où ils sont 40 %. La situation est particulièrement délicate dans le secteur hospitalier : en 2015, les accidents du travail ont touché 4 % des agents hospitaliers, le plus souvent à la suite d'efforts liés à la manutention des patients. Au départ, le Gouvernement souhaitait renvoyer l'ensemble du sujet à une ordonnance. La commission a préféré inscrire « en dur » certaines garanties en s'inspirant du rapport de Catherine Di Folco et de

du renforcement de la période de préparation au reclassement, de la mutualisation des médecins de prévention, du rendez-vous de carrière pour les métiers les plus pénibles. J'ajoute que, sur l'initiative de notre collègue Jocelyne Guidez, nous avons également étendu le congé de proche aidant à la fonction publique. Le texte de la commission permet donc des avancées rapides pour répondre à des problèmes concrets, alors que les ordonnances ne seront pas publiées avant douze à quinze mois. Enfin, mes chers collègues, nous vous demanderons le retrait de plusieurs de vos amendements qui nous semblent déjà satisfaits par le texte de la commission.

protection sociale complémentaire, de santé au travail, de temps partiel thérapeutique et de congés. Chacun de ces sujets, de notre point de vue, revêt une grande importance pour les agents publics. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le Parlement de s'en dessaisir, d'autant que les quelques orientations évoquées dans l'étude d'impact- fusion des instances médicales, restriction de la visite médicale à un certain type d'emplois -font craindre une moindre prise en compte des enjeux liés à la santé au travail.

Dans les cas du rendez-vous de carrière et du renforcement de la période préparatoire au reclassement, il s'agit de mieux prévenir les risques professionnels, en s'inspirant du rapport Di Folco-Marie.

pour dresser un état des lieux de la protection sociale complémentaire et des niveaux de participation des agents publics dans les trois versants de la fonction publique nous sera bientôt remis ; il sera également communiqué aux partenaires sociaux à l'occasion d'une réunion de travail organisée le 18 juillet. C'est sur la base de ce rapport

prochainement remises, nourriront cette concertation. J'aurai l'occasion de revenir sur un certain nombre de dispositions adoptées par la commission des lois, dont nous partageons l'objectif, même si nous considérons qu'elles sont peut-être de nature à préempter

Depuis le 1 janvier 2017, le centre de gestion du Rhône propose un nouveau service aux collectivités, le service de médecine statutaire et de contrôle, qui a pour objet de vérifier l'aptitude à l'embauche d'un candidat et de contrôler la justification médicale des arrêts de travail des agents. des agents. Assurée par un médecin agréé intégré au centre de gestion, cette mission est accessible par convention. Après plusieurs mois de fonctionnement, le centre de gestion a constaté une montée en charge progressive de l'activité opérationnelle, notamment de contrôle, et une baisse sensible de l'absentéisme. L'objet de cet amendement est de permettre le développement de cette mission, de manière sécurisée, dans l'ensemble des centres de gestion. Quel est l'avis de la commission ?

est à M. le secrétaire d'État. À la suite de mon propos de l'instant précédent, j'indique que le Gouvernement est favorable tant à la création du congé de proche aidant qu'à la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive dans les trois versants de la fonction publique. Cet amendement vise à conserver ces mesures adoptées en commission des lois tout en sécurisant les droits, s'agissant du congé des proches aidants. En revanche, nous ne souhaitons pas préempter la concertation à venir avec les organisations syndicales et les employeurs publics sur la question de la prévention de l'inaptitude et le maintien dans l'emploi. C'est pourquoi nous proposons la suppression

ont omis de faire référence à l'article L. 3142-26 du code du travail. Par ailleurs, le dispositif retenu fait expressément mention de l'article L. 3142-25-1 du même code. Premièrement, l'article L. 3142-25-1 du code du travail codifie l'article 1 de la loi du 13 février 2018 L'article 3 de cette loi prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de l'article 1 aux agents publics civils et militaires. Or ce décret a été pris, ce qui rend cette référence inutile. Deuxièmement, l'article L. 3142-26 du code du travail dispose que « pour mettre en oeuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise détermine : 1° La durée maximale du congé ; 2° Le nombre de renouvellements possibles ; 3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé 4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel. » En omettant de faire référence à cet article, l'actuelle duplication aux fonctionnaires des dispositions relatives au au congé de proche aidant n'est que partielle. En apportant une précision, les auteurs de cet amendement visent le même but que la commission. Considérant que l'article 1 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique permet que se tiennent des négociations entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers sur des sujets relatifs aux ressources humaines, rien ne fait obstacle à l'application de l'article L. 3142-26 aux agents publics, sous réserve des précisions relatives à la manière dont cet article doit être appliqué aux agents publics. En effet, cet amendement ouvre la possibilité- il ne s'agit pas d'une obligation -de négocier sur les conditions du congé de proche aidant. Enfin, l'amendement n° 440 rectifié déposé par le Gouvernement a permis de rendre recevable une précision complétant l'objectif de l'amendement.

Dans la fonction publique territoriale, plus de 76 % des agents sont de catégorie C, exerçant souvent des métiers à hauts facteurs de pénibilité. Cet amendement a pour objet d'instituer un bilan de carrièreau terme de dix années d'exercice, afin de prévenir des situations éventuelles d'inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l'usure physique, et d'examiner les possibilités d'évolution professionnelle ou de reclassement. Il a également pour objet de prévoir que, en dehors de la période de préparation au reclassement, un agent en disponibilité d'office pour raison de santé qui n'est pas définitivement inapte à tout emploi pourra exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Enfin, cet amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d'une période de préparation au reclassement, d'être mis à disposition par un centre de gestion auprès d'une autre collectivité.

Ce phénomène touche toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, et entraîne une augmentation des demandes de retraite pour invalidité ou des licenciements pour inaptitude. Notre amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d'une période de préparation au reclassement, d'être mis à disposition par un centre de gestion auprès d'une autre collectivité pour lui permettre ainsi d'être effectivement reclassé.

Ce sont ces mêmes agents qui sont exposés quotidiennement à des exigences professionnelles à hauts facteurs de pénibilité, leurs conditions matérielles de travail organisant inévitablement leur usure professionnelle.

d'inaptitude et d'examiner les possibilités d'évolution professionnelle. Ce bilan de carrière périodique compléterait l'entretien de carrière prévu à l'alinéa 24 du même article, qui vise à examiner les difficultés rencontrées par les agents occupant des emplois présentant des risques professionnels majeurs et à déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelle. Pour être tout à fait complet, j'indique qu'il est prévu que ce bilan soit assuré par l'autorité territoriale ou le centre de gestion, un décret en Conseil d'État déterminant les modalités d'application de cette disposition.

est à M. Arnaud de Belenet. Cet amendement vise les cas de disponibilité d'office pour raisons de santé, c'est-à-dire les cas où un agent n'est plus en capacité physique d'assurer ses missions. cas est un peu différent des précédents. Nous proposons d'ajouter une nouvelle voie aux solutions actuelles, qui ne sont pas pleinement satisfaisantes, en permettant à l'agent d'exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. L'avis du comité médical compétent serait alors évidemment requis. Dans le droit actuel, cette possibilité est réservée aux bénéficiaires d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Bien évidemment, nous ne pouvons pas sous-estimer l'effet positif d'une activité, même de faible importance, pour un agent qui serait confronté à une telle situation de mise en disponibilité d'office pour raisons de santé. Nous devons encourager la possibilité de maintenir un lien avec le travail et les missions de service public lorsque cela est médicalement possible.

de proche aidant, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 577 de la commission. Le Gouvernement souhaite en effet attendre pour régler les problèmes de santé au travail. Les conclusions du rapport de Mme Di Folco et de M. Marie, qui a fait l'objet d'une concertation avec toutes les parties prenantes, permettent toutefois d'avancer dès à présent. Nous demandons par conséquent le retrait de l'amendement n° 498 rectifié, qui nous paraît partiellement satisfait par l'amendement du Gouvernement. De même, il nous semble difficile de transposer les modes de négociation du secteur privé au secteur public. Nous demandons également le retrait des amendements identiques n 353 rectifié et 558 rectifié. Le texte de la commission prévoit d'ores et déjà l'organisation d'un bilan de carrière.

que la concertation autour de l'ordonnance prévue à l'article 17 permettra d'apporter des réponses sans qu'il soit nécessaire d'être aussi précis à ce stade dans la rédaction « en dur », pour reprendre une expression de M. le rapporteur.

: le Gouvernement n'est pas favorable à l'idée consistant à permettre à un agent en période de préparation au reclassement d'être mis à disposition par un centre de gestion auprès d'une autre collectivité pour exercer des missions temporaires de remplacement. Il nous semble nous semble plus opportun de veiller à préserver l'objectif même de la période préparatoire au reclassement, qui est d'accompagner les fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions vers un reclassement dans des postes en adéquation avec leur état de santé et leur projet professionnel. Les mises en situation professionnelle, dans le cadre de collectivités différentes, sont rendues possibles par les textes qui régissent la période préparatoire au reclassement sans qu'il soit nécessaire d'aller jusque vers des mises à disposition, qui nous paraissent être d'une autre nature.

n° 518, qui vise à permettre aux fonctionnaires mis en disponibilité d'office d'exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation, car il existe déjà dans notre droit des dispositions tendant à favoriser le maintien dans l'emploi des agents en situation d'inaptitude ou de congé maladie. Je pense ainsi à l'exercice d'une activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation ou au droit, que je viens d'évoquer, à une période de préparation au reclassement. Cette question se pose- et M. de Belenet l'a

En effet, l'exercice de la médecine du travail a été largement assoupli dans le régime général, et il me semble que la fonction publique territoriale a besoin que ces mesures d'assouplissement lui soient rapidement étendues pour favoriser la préservation des politiques de prévention de la santé au travail. Il est également proposé d'étendre l'application à la fonction publique des dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contrôle de l'absentéisme en cas d'incapacité au travail. travail. Les règles de contrôle de l'absentéisme dans la fonction publique territoriale relèvent de dispositions juridiques complexes, et il serait, à mon sens, cohérent et équitable que ces dispositifs de contrôle de l'absentéisme dans la fonction publique soient similaires à ceux du régime général, garantissant ainsi aux employeurs publics la mise en oeuvre d'un système expérimenté, incontestable et efficace dans la lutte contre l'absentéisme abusif au travail, dont on sait qu'il est malheureusement plus important dans la fonction publique que dans le secteur privé. Quel

Concernant l'absentéisme, la réintroduction du jour de carence commence à porter ses fruits dans la fonction publique, comme l'a démontré un récent rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale. L'économie est estimée à plus de 120 millions d'euros pour la seule année 2018. Concernant les médecins de prévention, la commission a proposé des mesures concrètes pour répondre à ce problème récurrent. Elle a renforcé la mutualisation des services de prévention et permis, à titre expérimental, à des médecins agréés d'exercer les fonctions de médecin de prévention. C'est donc une demande de retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

2007, a atteint 9,5 % en 2016 dans la fonction publique territoriale, contre à peine 4,6 % dans le privé, selon le baromètre Ayming. Ainsi, en 2017, la facture s'est élevée à 4 milliards d'euros, presque une fois et demie les économies annuelles demandées sous le quinquennat précédent. Cet amendement vise donc à rétablir une certaine justice sociale et financière en rémunérant les agents autorisés à travailler à temps partiel, en congé maladie ou maternité, en fonction de ce à quoi ils ont réellement droit.

Deuxièmement, les collectivités territoriales concluraient avec le centre de gestion auquel elles sont rattachées une convention d'accompagnement pour ces agents. En conséquence, cet amendement vise à prévoir, pour les centres de gestion, la compétence en matière d'employabilité dans l'objectif de mobilité professionnelle. Quel

En outre, la commission a déjà prévu un rendez-vous de carrière, à l'article 17 du projet de loi, pour mieux anticiper les reconversions professionnelles. Enfin, l'article 22 du présent texte habilite le Gouvernement

et les agents occupant des postes avec un risque d'usure professionnelle prononcé.

imputable à l'exercice militaire. Il s'agit de personnes qui ont achevé leur carrière militaire, qui ont fait l'objet d'une blessure dans le cadre de cet exercice militaire et qui, quelques mois ou quelques années après, du fait des conséquences de cette blessure, doivent interrompre la nouvelle activité qu'ils

pour toutes les autres décisions d'ordre individuel relatives à l'avancement ou à la promotion, il nous semble nécessaire de maintenir l'avis de la commission administrative paritaire pour les décisions d'avancement exceptionnel des policiers municipaux. En outre, contrairement au Gouvernement, nous estimons que les obligations de formation actuellement prévues par les statuts particuliers en cas d'accès à un cadre d'emploi supérieur ne seraient pas applicables en cas de promotion ou d'avancement à titre exceptionnel. Enfin, je réitère le rappel que j'ai formulé en commission : en

1225-16 du code du travail, complété par l'article 87 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, permet déjà à une salariée du secteur privé bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation, ainsi qu'à son conjoint, de bénéficier d'une autorisation d'absence. L'article 163 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté étendait ces dispositions aux agentes publiques, mais le Conseil constitutionnel les a censurées dans sa décision du 26 janvier 2017, pour des motifs de procédure. Ces situations ne nous semblent pas couvertes par la rédaction de l'article 17, lequel n'évoque que la parentalité. Nous proposons donc de préciser l'article 17 en ce sens.

Mme le rapporteur. Par souci de lisibilité et d'intelligibilité, cet amendement vise à toiletter les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

M. Didier Marie. Avec cet amendement, nous proposons d'aligner le régime des congés pour décès familial pour les trois versants de la fonction publique sur le régime, plus favorable, dont bénéficient les salariés relevant du code du travail. Ainsi, le congé en cas de décès d'un enfant serait porté à cinq jours, contre trois actuellement dans la fonction publique. En outre, les congés pour décès familiaux seraient élargis aux cas de décès des beaux-pères et belles-mères. Enfin, un congé familial de deux jours serait créé en cas de survenance d'un handicap chez un enfant. Dans chacune de ces hypothèses, le texte prévoit une durée minimale,

par le congé de solidarité familiale, qui peut être activé lorsque le pronostic vital d'un membre de la famille est engagé. De surcroît, la commission a créé « en dur » le congé de proche aidant, à l'article 17.

préalablement à la publication de ce décret, nous tenons à disposer d'un temps de concertation avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs publics, notamment territoriaux. En effet, un vrai travail d'harmonisation est nécessaire : de leur propre initiative, un certain nombre d'employeurs ont d'ores et déjà mis en place des autorisations spéciales d'absence.

présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes. Il introduit le droit de disposer d'une heure par jour afin d'allaiter son enfant, au besoin sur son lieu de travail, pour les fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique. Ce droit serait limité à la première année suivant la naissance du ou des enfants concernés. Pour l'heure, il nous semble qu'aucune disposition ne donne un tel droit aux mères travaillant dans la fonction publique. Nous comprenons donc difficilement l'amendement de suppression déposé par le Gouvernement, et nous émettons un avis défavorable. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Ce n'est là que la reprise du droit applicable aux salariés du secteur privé et, plus précisément, de l'article L. 1225-30 du code du travail. Pourquoi refuser la reconnaissance de ce droit aux agents publics ? L'objet de votre amendement, qui tient en deux phrases quelque peu sibyllines, avance qu'« il n'est pas nécessaire de créer un congé de la position d'activité ». Ce n'est toutefois pas le sens de notre article : nous créons simplement une autorisation d'absence d'une heure,

Une seule exception est prévue, lorsque l'administration possède « une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants ». Dès lors, les services « devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant vous en conviendrez -c'est rarement le cas, malheureusement. Cette interprétation a été confirmée par une réponse à une question écrite d'un sénateur, datée du 6 octobre 2016. Le Défenseur des droits a également regretté cette situation dans son rapport de 2018,

sonne comme une provocation pour l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, jetés en pâture à la vindicte populaire, suspectés d'être des tire-au-flanc alors que, le plus souvent, ils participent avec dévouement à l'exécution des services publics locaux, sans compter leur temps. Ainsi, cet article engage les collectivités à opérer une harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du travail, soit 1 607 heures annuelles. Pourtant, jusqu'à présent, l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 26 janvier 1984 prévoit que « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées

de définir et de choisir la durée de travail des agents, bien sûr dans le cadre légal, en ne pouvant infléchir cette durée que dans un sens favorable à ces agents. D'ores et déjà, cette faculté d'appliquer des temps de travail plus favorables est largement encadrée. Ainsi, le même article de la loi de 1984 prévoit la possibilité de maintenir des régimes inférieurs à la durée légale, à la double condition qu'ils aient été mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 2001 et que cette dérogation ait été formalisée par une décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité, après avis du comité technique. Selon l'étude d'impact, la durée annuelle de travail serait inférieure de moins de 30 heures à la durée légale. Pour 30 petites heures annuelles, est-ce bien sérieux d'obliger l'ensemble des collectivités à revoir leur régime de temps de travail ? N'ont-elles pas d'autres urgences à régler ? Est-ce le problème majeur affectant la qualité du service public local ? Nous ne le croyons pas. Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposerons la suppression de cet article provocateur, qui remet en cause la libre administration des collectivités territoriales et qui va se traduire par un recul des droits acquis pour les fonctionnaires territoriaux. La parole

Didier Marie, sur l'article. La question du temps de travail dans la fonction publique sert souvent de chiffon rouge pour dénigrer le fonctionnaire,

portait sur 1,1 million d'agents, parmi les 2,4 millions que compte la fonction publique de l'État. Il constatait que 310 000 agents travaillaient moins de 35 heures par semaine, dont 120 000 en raison de compensations liées à des sujétions inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

qui ont bénéficié d'un accord avant 2001 et ceux qui auraient fait l'objet de dispositions particulières après. Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, deux rapports sont aujourd'hui connus : celui de M. Philippe Laurent, qui atteste

En effet, si la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes invitent régulièrement les collectivités à contenir leurs charges de personnel en agissant sur les effectifs et le temps de travail, d'autres études sont éclairantes. Le rapport de la Dares, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, sur la fonction publique territoriale, ou celui du vice-président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, M. Philippe Laurent, publié en 2016 et toujours d'actualité, nous apprennent ainsi que près de la moitié des fonctionnaires de la fonction publique territoriale-

42 % des agents travaillent le samedi et 30 % le dimanche ; et que le temps de travail moyen, dans la fonction publique territoriale, atteint 1 637 heures par an, soit davantage que le temps légal annuel de 1 607 heures. Telle est la réalité des chiffres

si l'on se réfère à la durée légale retenue par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2016 sur les finances publiques locales- 1 562 heures -, la mesure proposée constituerait une économie globale de l'ordre de 1,2 1,2 milliard d'euros selon la juridiction financière. L'impact, en termes d'effectifs, d'un retour de l'ensemble des agents territoriaux aux 1 607 heures annuelles a été chiffré par la Cour des comptes à un gain de 57 000 équivalents temps plein, ou ETP.

tous à des situations spécifiques imposant des organisations de service très particulières, car les métiers de la fonction publique territoriale sont innombrables, avec des astreintes, du travail de nuit et du travail le week-end. Il s'agit donc d'un simple prétexte pour poursuivre la mise en oeuvre de votre plan de destruction de l'emploi public.

d'autre part, que la rédaction que nous avons proposée à l'Assemblée nationale permet d'écarter explicitement du champ de ce débat l'ensemble des personnels enseignants ou de recherche. Nous avons en outre indiqué à plusieurs reprises- comme certains d'entre vous

en effet un écart entre le contrat de travail, l'engagement, la durée du travail de l'agent et la réalisation effective ou non du temps de travail.

j'ai mis en oeuvre un certain nombre de dispositions pour réduire le nombre de jours de congé, qui ne paraissait pas justifié, et pour ouvrir la discussion sur l'annulation des congés d'ancienneté qui existaient dans ma collectivité, sans fondement légal. Ma successeur, auprès de qui je reste engagé comme conseiller municipal, a eu l'occasion de délibérer en mars 2018, mois suivant la communauté d'agglomération à laquelle j'ai la chance d'appartenir, pour revenir sur un accord antérieur à 2001 et ainsi, d'une certaine manière, appliquer avec quelques mois d'avance la disposition que je propose pour l'ensemble des collectivités.

se déroule dans un délai de douze mois, à compter non pas de la publication de la loi, mais du renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités concernées, c'est-à-dire douze mois après mars 2020 pour les communes et les intercommunalités et douze mois après le renouvellement de 2021 pour les régions et les départements.

est ainsi libellé : La parole est à Mme Sylviane Noël. L'article 18 permet une harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires, les collectivités territoriales disposant d'un délai d'un an à compter du prochain renouvellement des exécutifs locaux pour définir de nouvelles règles relatives au temps de travail des agents.

Le Gouvernement propose, par l'amendement n° 387, de ramener à douze mois le délai dont bénéficieront les employeurs publics territoriaux ayant maintenu des régimes dérogatoires pour redéfinir des règles de temps de travail conformes au droit commun.

que, en Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le collège des employeurs territoriaux, qui était favorable à une application des 35 heures, avait lui-même déposé un amendement pour que cette période puisse atteindre deux ans,

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement tend à préciser que les nouvelles règles relatives au temps de travail entrent en application le 1 janvier suivant la date à laquelle elles auront été définies par l'autorité territoriale, ce qui ne me paraît pas souhaitable. Pour les agents soumis à un cycle de travail correspondant à une année civile, il est évident que les nouvelles règles entreront pleinement en application au 1 janvier suivant, mais ce n'est pas le cas partout et pour tous les agents. La commission demande donc le retrait de cet amendement ;

L'article 18 oblige à renégocier les accords locaux sur le temps de travail conclus antérieurement à l'adoption de la norme des 1 607 heures annuelles dans les dix-huit mois qui suivent le renouvellement des assemblées. Dans sa rédaction actuelle, il fait l'impasse sur les raisons qui ont prévalu à la négociation de tels accords

l'avis de la commission ? Cet amendement vise à ce que les sujétions particulières auxquelles sont soumis certains agents territoriaux soient prises en compte dans la définition du temps de travail. est pleinement satisfait par la rédaction actuelle de l'article 7-1 de la loi statutaire et par le décret du 12 juillet 2001 pris pour son application. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

me vaudra pas que des amis ... Il porte en effet sur la définition hebdomadaire du service des enseignants du second degré, laquelle entraîne des rigidités dans le fonctionnement des établissements et a pour conséquence la perte d'un nombre appréciable d'heures d'enseignement pour les élèves.

aux besoins de l'institution et à l'intérêt des élèves. Il vise à définir les obligations de service des enseignants du second degré sur une base annuelle et non plus hebdomadaire, en tenant compte de la durée annuelle de travail effectif mentionnée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Les enseignants du second degré se trouveraient dès lors dans la même situation

Il correspond à une recommandation ancienne, reprise par nos collègues Max Brisson et Françoise Laborde dans leur récent rapport sur le métier d'enseignant. M. Brisson n'est pas de ceux qui entretiennent des fantasmes sur le temps de travail des enseignants ce n'est pas parce que les enseignants du secondaire assurent entre 15 et 20 heures de cours hebdomadaires qu'ils ne travaillent que 15 à 20 heures par semaine ; il faut évidemment ajouter le temps de préparation des cours, de correction des copies, de participation aux travaux des équipes pédagogiques, de permanence dans l'établissement. Nous le savons tous, comme nous savons que le métier d'enseignant est difficile et souvent éprouvant physiquement et mentalement. La représentation nationale se doit de le reconnaître et de témoigner sa confiance à l'égard de ces professionnels, qui jouent un rôle déterminant pour la formation de la jeunesse comme pour la cohésion de notre société. Nos professeurs sont d'ailleurs moins bien payés que la moyenne de l'OCDE et même deux fois moins bien qu'en Allemagne en début de carrière. L'annualisation des obligations de service, comme le soulignent nos collègues Brisson et Laborde, n'aurait pas pour objet de faire davantage travailler les enseignants, mais de mieux répartir leur temps de travail et de mieux tenir compte du temps de présence en établissement en dehors des cours. Elle pourrait également limiter les situations dans lesquelles un enseignant se trouve contraint de partager son service hebdomadaire

Contrairement à ce que vient d'exprimer Mme la rapporteur à l'instant, nous considérons que le maintien d'une norme hebdomadaire est un gage d'équité et d'organisation auquel le

d'expérimenter la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, sous réserve d'un accord majoritaire des enseignants, ce qui fait sauter un verrou supplémentaire. Nous avions exprimé nos inquiétudes quant à cette mesure. Cet amendement tend à aller encore plus loin en sortant du seul domaine de l'expérimentation pour ouvrir la porte à une annualisation des heures,

Cette mesure risque de dégrader profondément leurs conditions de travail. Elle n'est donc pas acceptable. Elle serait, surtout, préjudiciable pour les élèves, qu'elle se traduise par un changement d'enseignant en milieu d'année ou par un rythme d'apprentissage déséquilibré par le regroupement des heures de certaines matières sur des périodes plus courtes. Rien de tout cela n'est dans leur intérêt. Nos enfants ont besoin de stabilité et de régularité, le processus d'apprentissage nécessite de prendre du temps. L'étalement sur une année leur permet d'assimiler petit à petit le savoir qui leur est transmis ; l'alternance des matières rythme une journée, une semaine. C'est ainsi que l'on apprend, en reprenant ce qui a été vu au cours précédent, durant l'ensemble de l'année scolaire. Le cadre réglementaire du service des enseignants doit absolument être maintenu, car il s'agit d'un garde-fou essentiel pour préserver à la fois les conditions de travail des enseignants et celles des élèves.

M. Max Brisson, pour explication de vote.

remarques à propos de la pédagogie et des élèves. L'annualisation du temps de travail des enseignants est au service des élèves, dans la mesure où elle doit permettre une organisation pédagogique beaucoup plus souple et la construction de projets d'établissement.

que sur des bases déclaratives. Les organisations syndicales sont d'ailleurs fondées à parler de « travail caché », ce qui ne permet pas de bien valoriser la fonction enseignante. Voilà pourquoi, malgré le peu d'appétence de notre institution, de la commission des lois et particulièrement de son président, pour les rapports demandés au Gouvernement, cet amendement vise, dans un souci de bonne politique et de transparence, que le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport recensant le temps de travail effectif des professeurs du premier et du second degré. Quel est l'avis de la commission ? Sans surprise,

dans son article. C'est probablement un choix judicieux pour lui, au vu des derniers chiffres rendus publics par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, qui a dressé

intégrer les personnels à statut particulier ; je pense notamment aux militaires, qui connaissent aujourd'hui un surdéploiement atteignant tout de même cent quarante jours annuels hors du domicile.

Il ne nous a pas paru choquant que la durée hebdomadaire de travail des agents de l'État soit fixée dans la loi, sans préjudice d'éventuelles adaptations pour tenir compte de sujétions particulières. L'avis est donc défavorable.

secrétaire d'État. Il s'agit de rétablir la référence à la durée légale du travail telle que définie par le code du travail, pour des raisons d'équité avec le secteur privé. Par ailleurs, nous proposons de supprimer la référence aux heures supplémentaires, qui, selon nous, pourrait être source de confusion dans l'application de la durée effective du travail.

au code du travail pour la détermination de la durée de travail hebdomadaire, tout en inscrivant dans le « dur » de la loi statutaire la base annuelle de décompte de 1 607 heures. Si l'on retenait la rédaction du Gouvernement, il faudrait modifier la loi statutaire le jour où l'on modifierait la durée hebdomadaire de travail dans le secteur privé.

qui, depuis 2017, ne précise plus que le télétravail doit être effectué de manière régulière. Faute de précision dans la loi, le décret a restreint les possibilités de télétravail à une organisation régulière

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à assouplir les dispositions légales relatives au télétravail dans la fonction publique, afin d'autoriser le passage ponctuel au télétravail, sur décision de l'employeur public et à la demande de l'agent. Cette proposition est cohérente avec les modifications apportées au régime de télétravail dans le secteur privé par l'ordonnance du 22 septembre 2017. La commission est donc favorable à l'amendement, d'autant que le télétravail, s'il est organisé convenablement et d'un commun accord entre l'employeur et l'agent,

les auteurs de cet amendement proposent que le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation conclu par les centres de gestion au niveau régional ou interrégional prévoie notamment l'incidence prévisionnelle de la mutualisation sur les effectifs des centres de gestion concernés et sur leurs dépenses de fonctionnement. Cet ajout nous semble superflu : la coordination, la mutualisation et la spécialisation ont bien pour objet, notamment, de dégager des économies d'échelle. second lieu, il est proposé que le schéma soit transmis pour avis au conseil d'administration de chaque centre. Cela nous semble impossible, puisque les centres de gestion sont les autorités décisionnaires en la matière : dans la mesure où ils approuvent le schéma, ils ne peuvent pas en

Nous n'avons pas modifié les conditions de majorité requises pour s'opposer au retrait, soit les deux tiers des employeurs affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou les trois les trois quarts des employeurs représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires. En revanche, nous avons prévu que, si les collectivités territoriales et établissements affiliés ne se prononcent pas dans un délai de trois mois, leur avis sera réputé défavorable. Ce dispositif nous paraît garantir un bon équilibre entre la liberté des collectivités territoriales volontairement affiliées et la nécessité de protéger les centres de gestion contre les décisions de retrait abrupt susceptibles de les déstabiliser fortement. L'avis est donc défavorable.

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif. Organisés sur une base départementale, ils sont chargés d'assister les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la gestion de leurs ressources humaines. Leurs missions ne sont pas mineures, puisque ces centres assurent notamment la publicité des listes d'aptitude et des créations et vacances d'emploi. Ils sont également en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, ainsi que du reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Autant de missions qui nécessitent proximité et dialogue permanent.

Nous ne sommes pas dupes : ces possibilités de fusion sont décidées selon des considérations uniquement budgétaires, puisqu'une fusion ne permet ni d'augmenter ni de mutualiser les moyens.

vise à permettre le transfert de plein droit des agents des centres de gestion qui décideraient de fusionner au centre de gestion issu de la fusion.

la commission n'y est pas favorable. La fusion librement consentie par les centres de gestion, c'est-à-dire par les collectivités et établissements adhérents, peut être un moyen d'améliorer le service rendu aux employeurs publics territoriaux comme aux agents. Le principe de mutualisation

elle n'a pas jugé opportun de donner compétence à la conférence régionale de l'emploi et de la formation pour dresser et réviser le bilan du schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation établi par les centres de gestion. Je rappelle que ce schéma remplacera les chartes élaborées par les centres qui décident d'organiser des missions au niveau régional. Nous avons à cet égard un léger désaccord de fond. Il faut bien se représenter que cette présentation va de pair avec l'obligation prévue par le projet de loi d'établir ce schéma au niveau régional. Quoi de mieux, en l'espèce, que de soutenir l'effort de mutualisation et de spécialisation

pour coordonner les missions des collectivités territoriales et des centres de gestion. Il me paraît cohérent que le bilan des schémas de coordination se fasse au sein des conférences régionales, chargées de la coordination des missions en matière d'emploi public territorial. Quel est l'avis de la commission ? l'avis de la commission ? Il n'appartient pas à la conférence régionale de l'emploi d'établir un bilan du schéma de coordination conclu par les centres de gestion, encore moins de le réviser. Par ailleurs, on ne voit pas comment, en droit,

est à Mme Sylviane Noël. Dans le cadre de leur mission d'information sur l'emploi public territorial, les centres de gestion sont chargés d'établir un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ils ont également compétence pour la collecte des données sociales en vue de l'élaboration du rapport sur l'état de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du service, au travers des bilans sociaux présentés par l'autorité territoriale au comité technique. C'est ainsi que les centres de gestion ont pu, lors de leur dernière campagne de recueil de données, collecter les données sociales relatives à près de 1,5 million d'agents de la fonction publique territoriale.

de la loi du 26 janvier 1984 communiquent au centre de gestion de leur ressort les informations constitutives du bilan social. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement